a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Louis Moinard, qui fut sénateur de la Vendée de 1987 à 2004. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 16 , alinéa 2 du règlement, la proposition de création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique

Les préfectures sont chargées du travail de recensement de la voirie de l'ensemble des communes. Toutefois, celui-ci se fait sur une base déclarative : il appartient aux conseils municipaux de délibérer pour classer ou déclasser dans le domaine public communal les voies désignées et de transmettre aux préfectures leurs délibérations. Les préfectures informent ensuite chaque année la DGCL des modifications des linéaires de voirie communale ainsi recensées, afin que ces variations puissent être prises en compte pour le calcul de la dotation de solidarité rurale. L'État publie chaque année les données utilisées pour le calcul de la DGF en format ouvert et réutilisable, y compris l'ensemble des longueurs de voirie déclarées chaque année. La parole

ne permet pas aux agents de bénéficier de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation déplafonnée, comme ils pourraient y prétendre en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2008. Ce texte prévoit qu'une prime déplafonnée s'applique lorsque le service a la charge de voies sous tunnel de plus d'un kilomètre. Or le CEI de Murat entre parfaitement dans ce cadre, puisque les agents assurent l'exploitation et l'entretien du tunnel du Lioran, long de plus de 1 500 mètres, soit 50 % de plus que la longueur minimale

Le rôle de ce tunnel est donc stratégique pour éviter un col de montagne particulièrement sinueux et difficile. En outre, lorsqu'un incident se produit à l'intérieur du tunnel, comme cela arrive parfois, les agents du CEI de Murat doivent assurer la gestion du trafic routier par ce col, situé au coeur de la station de ski, ce qui constitue une difficulté et une responsabilité supplémentaires, notamment en raison de l'affluence de milliers de skieurs et de visiteurs.

Leur engagement mérite respect et considération. Cinq accidents mortels ont malheureusement eu lieu depuis 2020, ce qui nous rappelle cruellement à quel point ce métier est à la fois crucial et trop souvent dangereux. Comme vous le soulignez, le décret du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement précise que cette gratification « est fixée au sein de chaque service par type de postes de travail homogène en tenant compte des contraintes [ ...], notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches, ainsi que de la technicité des missions Il précise également que les « agents [ ...] affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal Ces postes sont notamment ceux qui sont liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à la gestion des tunnels routiers. Le centre d'entretien et d'intervention de Murat est donc bien éligible au déplafonnement du montant maximal de la prime, et les agents affectés dans ce centre bénéficient aujourd'hui d'un montant de prime déplafonné, c'est-à-dire supérieur à deux fois le montant minimal fixé par l'arrêté du 16 avril 2002, sans atteindre, comme vous l'indiquez à juste raison, les montants maximaux figurant au b de l'article 2 de l'arrêté susmentionné. Toutefois, une révision du classement des centres est prévue dans le courant de l'année 2023, pour tenir compte des évolutions des contraintes d'exploitation. Dans ce cadre, le classement du centre de Murat fera l'objet

Le triage, tel qu'il a lieu pour l'instant, ne pourra donc plus se faire. Précisons que cette suppression est motivée par le fait que la gare est située sur le tracé des accès au tunnel du Lyon-Turin en projet.

le projet Lyon-Turin ne permettra pas de rattraper cette perte de report modal, car les porteurs du projet ont décidé que la Maurienne ne serait qu'un point de transit et de passage. C'est nier que son potentiel pourrait largement être développé grâce à l'industrie présente dans ce territoire. le ministre, ma question porte donc sur la pertinence et l'urgence d'une telle décision, anticipée en 2023 pour une mise en service théorique des accès français du Lyon-Turin après 2040- pour ne pas dire aux calendes grecques

je comprends votre inquiétude face à la fermeture du site de Saint-Jean-de-Maurienne. Le Gouvernement est pleinement engagé pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de décarbonation, et le soutien au rail en est l'une des composantes essentielles. Comme vous l'avez souligné, cette fermeture est liée au projet Lyon-Turin, plus spécifiquement au raccordement du nouveau tunnel de base au réseau ferré national à Saint-Jean-de-Maurienne. Celui-ci nécessite la construction d'ouvrages occupant toutes les emprises ferroviaires de la gare, dont les voies de service que vous évoquez. Le déménagement de l'activité de fret, basculée vers Saint-Avre, a été préparé depuis 2015 entre SNCF Réseau et Fret SNCF, qui est le seul utilisateur du site. La capacité disponible en gare de Saint-Avre a été dimensionnée en conséquence pour absorber le trafic existant, mais d'éventuels besoins complémentaires pourraient également être traités en mobilisant des voies disponibles sur d'autres sites de la ligne. Le projet Lyon-Turin a notamment pour objectif de permettre un report modal significatif du trafic transalpin des poids lourds vers le rail. Il est donc positif pour le développement du fret ferroviaire, un secteur pour lequel nous allons renforcer le soutien public. Comme le ministre délégué chargé des transports l'a annoncé cette semaine, l'État augmentera ainsi de 30 millions d'euros le montant des aides à l'exploitation à partir de 2025 et ce jusqu'en 2030, portant le tout à près de 330 millions d'euros, contre moins de 100 millions d'euros avant 2020.

et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Monsieur le ministre, les récentes déclarations du ministre Clément Beaune laissent entrevoir la possibilité d'une réduction de la part des projets routiers, pour donner une priorité aux transports publics et aux transports ferroviaires. À cet effet, une étude d'opportunité environnementale a semble-t-il été programmée pour donner d'ici à l'été prochain un nouvel avis sur une cinquantaine de projets d'infrastructures. Sept projets autoroutiers en cours sont concernés par ce réexamen,

dont la mise en concession a été lancée il y a un an et demi par Jean Castex, est parfaitement structurant pour le département d'Eure-et-Loir, notamment pour les communautés d'agglomération du Pays de Dreux et de Chartres métropole. Il doit maintenant voir le jour, d'autant que le choix du concessionnaire

le soutien à l'économie agricole et contribuera à l'amélioration de la sécurité et du cadre de vie des habitants en déviant le trafic de transit des zones urbanisées, ce qui réduira les nuisances et la congestion en entrée et en traversée d'agglomération. Je vous confirme que cette liaison fait pleinement partie de la revue des projets autoroutiers en cours. Cet exercice vise à réexaminer avec soin l'ensemble des projets à l'aune d'une série de critères dont le choix est plus que en particulier au regard de leur cohérence avec les engagements environnementaux du Gouvernement. Il s'agit également de tenir compte des spécificités locales et des bénéfices attendus de la réalisation de ces infrastructures, notamment en matière de désenclavement et de développement des territoires ruraux.

En effet, en application du code de l'urbanisme, l'opérateur qui souhaite réaliser un programme dans un tel secteur est tenu de joindre à sa demande de permis de construire un tableau indiquant clairement les surfaces planchers des logements créés au regard de ce qui est imposé par le plan local d'urbanisme Ainsi, l'obligation inscrite dans un PLU d'atteindre un seuil minimal de logements sociaux est bien vérifiée lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme, ce qui donne à cette règle son plein effet.

centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) en Île-de-France, afin d'accueillir le personnel oeuvrant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette mesure, si elle était mise en place, affecterait plus de 3 000 logements étudiants, qui seraient mobilisés pendant les mois de juillet et d'août 2024. La nouvelle de cette réquisition a créé une onde de choc parmi les étudiants, en particulier ceux qui avaient prévu de rester en région parisienne pendant cette période pour des raisons professionnelles ou personnelles. Les préoccupations soulevées sont multiples. Bien que le Crous ait affirmé que les étudiants concernés seraient relogés et exemptés de loyer pendant cette période, avec la garantie de retrouver leur logement à la rentrée, les organisations étudiantes ont exprimé des doutes quant à la capacité de cet organisme à honorer ses engagements sans créer de désagréments pour les résidents des établissements. En tant qu'élus, il est crucial que nous prenions cette situation au sérieux et fassions tout notre possible pour protéger les droits et le bien-être des étudiants. Par conséquent, monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les réquisitions de logements du Crous pendant les jeux Olympiques de Paris 2024. Les interrogations sont nombreuses et légitimes. Pouvez-vous confirmer ou infirmer ces informations qui préoccupent tant les étudiants ? En outre, si cette mesure devait être confirmée, il serait essentiel que le Gouvernement mette en place des mesures d'accompagnement solides, afin de minimiser les nuisances pour les étudiants et de garantir leur relogement adéquat.

En Île-de-France, plus de 7 000 hébergements Crous sont ainsi libérés chaque année entre les mois de juin et de septembre. Pour prendre part aux côtés des autres opérateurs à l'effort collectif pour le succès des jeux Olympiques et Paralympiques, le

bénéficieront exceptionnellement de la garantie de pouvoir récupérer un logement à la rentrée suivante, dès le 1 septembre. Pour les nouveaux habitants, les règles sont connues dès à présent : les douze résidences concernées ont une mention spéciale sur le site de candidature à un logement Crous.

6 000 l'année dernière, soit le double d'il y a dix ans -, qui suit le rythme de la croissance démographique exponentielle de la population guyanaise. Il s'agit aussi et surtout d'une demande unanime, légitimée par un réel besoin de prise en compte des problèmes spécifiques des étudiants de l'université de Guyane, qui n'est pas satisfait aujourd'hui, avec une gouvernance installée en Guadeloupe, au sein de laquelle la Guyane est faiblement représentée. au conseil d'administration du Crous Antilles-Guyane, la collectivité territoriale de Guyane n'est présente qu'un an sur trois, et, sur les sept représentants étudiants, un seul est élu de Guyane. En conséquence, les problèmes des étudiants guyanais, loin d'être ceux des étudiants antillais, sont peu abordés, Avec un PIB par habitant de 16 000 euros en Guyane, contre 25 000 euros aux Antilles, et un niveau de précarité plus grand, nos étudiants guyanais sont pourtant plus demandeurs d'aides sociales et d'accompagnement.

l'expression du Gouvernement est claire et constante : nous voulons allouer des moyens supplémentaires au bénéfice des étudiants guyanais. En revanche, il n'a jamais été question de créer de nouvelles structures administratives, dont le coût de fonctionnement ne serait pas corrélé corrélé à un niveau d'évolution positive pour les usagers. Sur la base de ces orientations, le service social de Guyane a été renforcé par une seconde assistante sociale.

En outre, une commission d'aide ponctuelle se réunit chaque semaine pour allouer des moyens aux étudiants les plus en difficulté. S'agissant des logements qui seraient en nombre insuffisant, il convient de relever que la résidence universitaire de aujourd'hui de nombreux logements vacants, dès le début de l'année scolaire. Quant à leur entretien, un programme de rénovation a pu être engagé et des améliorations ont été apportées, afin de mieux équiper les locaux et de renforcer le confort auquel les étudiants

Quant à la restauration universitaire à Cayenne, il est vrai que des malfaçons entravent malheureusement le bon fonctionnement du service de cuisine depuis la livraison du nouveau bâtiment.

reconnu par les lois de la République depuis 2011. Vous le savez, c'est une spécificité locale issue de l'histoire de ces départements et inscrite dans le code général de la fonction publique. Or l'application, à compter du 1 janvier 2022, de l'annualisation du temps de travail des agents de la fonction publique territoriale,

En effet, demander aux agents d'Alsace-Moselle d'effectuer le même nombre d'heures de travail que dans les autres départements revient à leur faire récupérer les heures correspondant aux deux jours fériés supplémentaires. Monsieur le ministre, de très nombreuses voix se sont élevées pour alerter le Gouvernement sur cette méconnaissance du droit local, qui n'a donné lieu à aucune concertation. Je me fais ici l'écho des nombreuses communes alsaciennes qui ont voté des motions et des délibérations pour qu'il soit tenu compte du droit local d'Alsace-Moselle et que soit respectée la durée annuelle de travail de leurs agents, soit 1 593 heures. Depuis le mois dernier, nous sommes également très nombreux à avoir signé la pétition du Conseil représentatif pour le droit local alsacien-mosellan pour s'opposer à la suppression des jours fériés, en soutien à notre droit local. L'interprétation qui est faite de cette annualisation constitue une menace réelle et inacceptable pour le droit local, auquel les Alsaciens sont fortement attachés. Par conséquent, ma question est très simple, monsieur le ministre : pouvez-vous nous confirmer, ainsi qu'aux collectivités locales d'Alsace-Moselle, que la loi de 2019 ne modifie en rien les dispositions du droit local ? La parole

afin d'harmoniser la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, mais également avec la fonction publique de l'État, l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique a supprimé les régimes de travail dérogatoires mis en place avant 2001 dans les collectivités territoriales. En vertu de cet article 47, les collectivités territoriales concernées étaient tenues de définir, dans un délai d'un an à compter du renouvellement général de leur assemblée délibérante, de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents. Cet article concerne évidemment les collectivités de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui se voient, par conséquent, appliquer la durée légale annuelle de travail effectif de 1 607 heures. L'article 3134-13 du code du travail prévoit, comme vous le rappelez, que dans ces départements le Vendredi saint et le 26 décembre sont des jours chômés. ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des 1 607 heures dans ces collectivités. La durée légale de travail s'applique, en effet, uniformément et indépendamment du nombre de jours chômés, qu'il s'agisse de jours fériés de droit commun ou des jours chômés propres aux départements de l'Alsace et de la Moselle. les collectivités territoriales et les établissements publics de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sauraient se prévaloir des deux jours chômés évoqués pour définir une durée annuelle de travail inférieure à 1 607 heures sans méconnaître les dispositions applicables en la matière.

de la fonction publiques. Monsieur le ministre, le métier de secrétaire de mairie est indispensable au fonctionnement de nos communes rurales. Les femmes et les hommes qui occupent cette fonction doivent être polyvalents, réactifs et répondre à des exigences d'expertise de plus en plus fortes. Aujourd'hui, nombre de maires de petites communes ont des difficultés à pourvoir ces emplois. Qu'en sera-t-il demain au regard des nombreux départs à la retraite attendus ?

Jusqu'à récemment, il collaborait avec Pôle emploi pour améliorer l'accès à ces formations. La participation financière de Pôle emploi permettait ainsi d'organiser une à deux sessions de formation de secrétaire de mairie par an. Le désengagement de Pôle emploi remet en question ces formations, alors même qu'elles sont grandement appréciées par les maires, les élus municipaux, les agents territoriaux et les demandeurs d'emploi. Je souhaiterais donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour consolider la participation financière de Pôle emploi, indispensable au maintien de ces formations. La parole

souhaitant rejoindre son service « Missions temporaires ». Cela se fait dans le cadre de la mission facultative de mise à disposition d'agents territoriaux, prévue à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, un centre de gestion à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local. Cette formation de vingt-neuf jours se décline en une partie théorique et en un stage pratique. Le CNFPT organise une formation théorique de quinze jours dans les domaines d'intervention des agents occupant l'emploi, ô combien essentiel, de secrétaire de mairie, comme l'état civil, l'urbanisme ou l'initiation à la commande publique. Le centre de gestion trouve un lieu de stage au sein d'une mairie du département, où le demandeur d'emploi sera encadré par un tuteur. De telles formations sont mises en oeuvre par plusieurs centres de gestion avec Pôle emploi, le CNFPT, les régions et d'autres acteurs locaux. La Fédération nationale des centres de gestion indique que le taux de retour à l'emploi à la suite de ces formations est de 90 %. Ces actions contribuent donc à renforcer l'attractivité de l'emploi de secrétaire de mairie et au retour à l'emploi de personnes au chômage. Les centres de gestion n'étant pas des organismes de formation, se pose la question du financement de ces formations. Des discussions sont actuellement menées, sous l'égide du cabinet du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

la ministre de la culture. Monsieur le ministre, dans le cadre de leurs projets d'aménagement, les collectivités doivent procéder à des fouilles archéologiques préventives. Conformément à la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, ces dispositifs visent à concilier la recherche scientifique, la conservation du patrimoine et le développement socioéconomique. Cependant, nous constatons que les plus petites collectivités sont souvent confrontées à des coûts dépassant largement leurs capacités financières. Par conséquent, elles sont contraintes d'abandonner leurs projets et de renoncer à leurs ambitions en matière de développement territorial. Bien que le Fonds national pour l'archéologie préventive ait été mis en place pour subventionner les opérations de fouilles archéologiques, dont le coût pourrait compromettre l'équilibre financier des projets d'aménagement, les critères d'éligibilité actuels rendent son accès difficile- voire impossible -pour de nombreuses collectivités. Dans ce contexte, il est essentiel d'envisager l'élargissement du périmètre des subventions, afin de répondre aux besoins des collectivités. En outre, la mutualisation des dépenses contribuerait également à mieux accompagner ces plans d'aménagement. Ainsi, je souhaiterais savoir comment le Gouvernement prévoit de soutenir financièrement les collectivités, en particulier les petites communes, afin de surmonter ces difficultés. Il est primordial que nous travaillions ensemble pour trouver des solutions et garantir que toutes les collectivités,

La parole est à M. le ministre délégué. Monsieur le sénateur François Bonneau, la France a mis en place un dispositif d'archéologie préventive visant à concilier les exigences de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social de nos territoires. Lors de l'instruction des projets d'aménagement, les services de l'État chargés de l'archéologie sont amenés à prendre des mesures permettant la détection et la sauvegarde, par l'étude, du patrimoine archéologique ou en garantissant sa préservation.

Le financement des fouilles repose essentiellement sur les maîtres d'ouvrage, sur la base de prix établis par les opérateurs présents sur le marché. Cependant, les aménageurs peuvent bénéficier d'aides financières, sous la forme de prises en charge ou de subventions, attribuées par le Fonds national pour l'archéologie préventive que vous avez mentionné,

L'archéologie préventive dispose donc d'un cadre juridique et financier adapté. Elle participe au développement de la politique culturelle, patrimoniale et scientifique soutenue par le ministère de la culture, tout en garantissant un aménagement raisonné du territoire, notamment en milieu rural. La parole

Première filière industrielle d'économie circulaire dans les territoires, renouvelable et à 100 % locale, la production de biogaz répond à l'ambition d'autonomie énergétique de la France et pourrait ainsi servir largement la décarbonation de la mobilité lourde. Pourtant, cette dynamique est en panne.

Prendre le pari de sortir des énergies fossiles, sans renforcer notre autonomie énergétique et notre avance technologique, constituerait une erreur de prospective majeure. Aussi mes questions sont-elles simples. Premièrement, le Gouvernement, qui a aussi limité ses soutiens au rétrofit électrique et hydrogène, entend-il, dans le cadre du plan d'action national en faveur du rétrofit récemment annoncé,

non seulement pour atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi pour en limiter les effets sur l'environnement, la qualité de l'air et la santé. En France, ce secteur est la première source d'émissions de gaz à effet de serre, avec 138 millions de tonnes équivalent CO2 émis en 2021.

en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. L'objectif de cette révision est d'accélérer la décarbonation du transport routier en cohérence avec les objectifs climatiques rehaussés de l'Union européenne, à savoir réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 d'ici à 2030, puis atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les négociations sur le projet de texte n'en sont encore qu'à leur début. La proposition de la Commission européenne prévoit des objectifs de réduction des émissions moyennes de CO2 à l'échappement des véhicules lourds neufs immatriculés au sein de l'Union européenne. Le choix des technologies pour atteindre ces objectifs appartient, en revanche, au constructeur. La proposition de révision du règlement prévoit également un objectif de 100 % de bus urbains neufs zéro émission, incluant les véhicules électriques à batteries, à pile à combustible et à hydrogène thermique. Par ailleurs, sur le plan national, comme il s'y est engagé le 13 avril dernier, le Gouvernement apportera un soutien de l'ordre de 100 millions d'euros en faveur de la trajectoire de décarbonation des transports lourds. La parole

De façon schématique, les collectivités dites « gagnantes », au regard du panier de recettes fiscales issues de la réforme, sont prélevées au titre du FNGIR au profit des collectivités dites « perdantes Les prélèvements et reversements au titre du FNGIR sont figés et reconduits chaque année pour un montant identique, ... Pourquoi ? ... en raison de la neutralité financière de l'époque. J'attire votre attention sur le fait que, dans la majorité des cas, payer le FNGIR est un avantage pour les communes. Cela signifie qu'elles ont reçu plus

Or ces ressources fiscales de compensation ont très souvent augmenté depuis 2011, alors que le prélèvement au titre du FNGIR est resté, quant à lui, figé.

Pour répondre à ces cas de figure, le Gouvernement a institué, dans la loi de finances pour 2021, un prélèvement sur recettes permettant aux communes ayant subi une perte de base de fiscalité économique de plus de 70 % depuis 2012 et pour lesquelles le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes de fonctionnement, de disposer annuellement d'une dotation de l'État à hauteur d'un tiers de leur prélèvement. Au titre de 2022, quelque 273 communes sont éligibles à cette dotation, pour un montant total de 246 millions d'euros.

Monsieur le ministre, j'ai récemment rencontré les syndicats de police de mon département, lesquels m'ont dressé un constat assez inquiétant. Aussi, permettez-moi de vous faire une synthèse de l'état des lieux. Si l'on prend l'exemple de la ville de Vierzon, celle-ci n'est pas dotée et risque de ne plus avoir de groupe de sécurité de proximité (GSP). De surcroît, cette commune ne dispose plus d'officiers. À Bourges, on observe trois départs pour une seule arrivée à l'occasion des mouvements dits « profilés

et de la gendarmerie, recrutement de plus de 7 000 policiers et gendarmes supplémentaires, création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, etc. En ce qui concerne le

La circonscription de sécurité publique de Vierzon s'appuie, pour sa part, sur un effectif opérationnel de 50 gradés et gardiens de la paix, soit un chiffre stable par rapport à la fin de 2016, mais en hausse par rapport à la fin de 2020. Nous allons être très attentifs à la situation de ce département, et je vous confirme que notre objectif est d'affecter douze policiers supplémentaires dans ces deux circonscriptions

Dans le Cher, comme partout en France, notre volonté est claire : déployer davantage de forces de l'ordre sur le terrain pour faire reculer la délinquance et répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens et de leurs représentants. La parole

Pour une commune de près de 3 000 habitants, le conseil municipal dénombre vingt-trois membres, soit un élu pour 130 habitants. À titre de comparaison, une ville d'environ 117 000 habitants, comme Besançon, chef-lieu de mon très beau département du Doubs, compte cinquante-cinq conseillers municipaux, soit un élu pour 2 127 habitants. Il est donc plus aisé de constituer une équipe municipale dans une grande ville que dans une petite commune rurale,

peu motivées. En résultent parfois un absentéisme non négligeable, voire des vagues de démissions quelque temps après l'élection. Le scrutin de liste, réservé aux communes de plus 1 000 habitants depuis la loi de 2013, complexifie encore davantage le recrutement de candidates et de candidats volontaires. Au regard de ces éléments, et forts de leur expérience personnelle, plusieurs maires de mon département, dont celle du Russey, souhaitent ouvrir une réflexion sur la possibilité de réduire le nombre de conseillers municipaux dans les plus petites communes. D'après eux, une telle évolution ne dégraderait pas la vie démocratique locale. Elle pourrait même l'améliorer, à condition que l'on renforce la formation des élus ; ces derniers seraient certes moins nombreux, mais mieux armés. cette mesure ne dégraderait pas non plus la qualité du lien entre les membres du conseil municipal et la population : le numérique constitue aujourd'hui un outil relationnel à même de compenser une légère réduction des équipes.

de participation à la vie publique tout en assurant le bon fonctionnement des conseils municipaux. Le législateur a tenu compte des difficultés que peuvent connaître les communes les moins peuplées pour trouver des candidats aux élections. Ainsi, en 2013, il a abaissé de sept à cinq le nombre de conseillers municipaux pour les communes de moins

au moins cinq membres dans les communes de moins de 100 habitants et au moins neuf membres dans les communes de 100 à 499 habitants.

intercommunale (EPCI), ainsi qu'au propriétaire et au titulaire d'un droit d'usage sur le terrain, de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. telle mise en demeure n'est possible que si la présence constatée viole les dispositions d'un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains dédiés. Par ailleurs, l'édiction d'un arrêté d'interdiction de stationnement, alors même que la commune ou l'EPCI ne remplit pas les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, est autorisée par la loi, notamment lorsque l'EPCI dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet.

l'opportunité de sa généralisation. La commission des délits et incivilités cités par des personnes ayant un mode de vie itinérant ne constitue pas, en soi, une dérive sectaire.

il convient de saisir le procureur de la République. Pour ce qui concerne les délits dénoncés et les dangers potentiels encourus par les enfants, il revient aux élus de procéder à des signalements au procureur de la République ou aux cellules de recueil des informations préoccupantes, qui relèvent des conseils départementaux. je vous remercie

repose sur le principe de l'imposition par l'État qui verse les revenus. Dès lors, les résidents français travaillant dans le secteur public belge seraient désormais imposés en Belgique, où le taux appliqué est bien plus élevé.

Par ailleurs, le statut dérogatoire des anciens frontaliers salariés du privé prendra fin dans une dizaine d'années. Ne serait-il pas judicieux de négocier dès maintenant le nouveau statut général des frontaliers ? Et ne pourrait-on pas, au passage, négocier un accord sur le télétravail ?

la nouvelle convention clarifiera le traitement fiscal des rémunérations de source publique. Elle repose, sauf exception, sur le principe de l'imposition par l'État qui verse ces revenus. Il s'agit là d'un choix logique, car ces revenus publics sont financés par les ressources publiques. Sur ce sujet, la rédaction de la convention signée par la France et la Belgique est conforme au modèle de l'OCDE. De telles dispositions se retrouvent couramment dans notre réseau conventionnel, en particulier dans les conventions négociées récemment. Cette nouvelle règle clarifie en réalité la situation des personnes qui perçoivent des rémunérations de source publique. Sur ce point, la convention n'entraîne des changements que pour une seule catégorie de travailleurs : les résidents français possédant la seule nationalité française, percevant des traitements publics de source belge

Le taux moyen des livrets ordinaires, fixé librement par les établissements bancaires, s'élevait quant à lui à 0,5 % en mars 2023. Comparés aux produits d'épargne réglementée des autres pays européens,

de collecte historiques. Notons aussi que la variation du taux du livret A a un impact sur d'autres acteurs que les épargnants, en particulier les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales. Leur dette contractée auprès de la Caisse des dépôts

le livret d'épargne populaire (LEP). Près de la moitié des Français sont éligibles à ce livret, dont le taux s'établit aujourd'hui à 6,1 %. Le Gouvernement a mené plusieurs actions de simplification et de promotion

l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays ». À ce titre, la Caisse des dépôts « est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite ». Placée « sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative », « elle est organisée par décret en Conseil d'État, pris sur la proposition de la commission de surveillance ». Le 9 février dernier, le journal annonçait en exclusivité

2021, la Caisse des dépôts a affecté quelque 170 milliards d'euros au financement du logement social et de la politique de la ville. Ces crédits ont permis de construire et de réhabiliter plus de 160 000 logements sociaux.

Sur 12,8 milliards d'euros de prêts versés par le fonds d'épargne en 2022, quelque 11,2 milliards d'euros, soit une part de 88 %, ont été consacrés au logement social et à la politique de la ville. À son bilan, le fonds d'épargne détient un encours de prêts au logement social de 174 milliards d'euros sur un total de 195,9

d'épargne finance d'ores et déjà d'autres projets d'intérêt général, quand le financement privé n'existe pas ou quand il se révèle insuffisant. C'est notamment le cas de projets menés par le secteur public local ; ils bénéficient d'une enveloppe de 28 milliards d'euros de prêts, ouverte jusqu'en 2027. Afin de rémunérer son passif, à savoir l'épargne réglementée des particuliers, le fonds d'épargne doit dégager du rendement sur ses actifs. La recherche de cet équilibre suppose d'obtenir un rendement moyen supérieur au coût de sa ressource. Dans un contexte de forte collecte et de taux élevé du livret A, cet enjeu revêt une acuité particulière. il est à la fois de bonne gestion et opportun pour le secteur HLM de diversifier les emplois du fonds d'épargne, précisément pour préserver son équilibre financier. En résumé, il existe aujourd'hui bien plus de liquidités disponibles sur le fonds d'épargne que de besoins de prêts à accorder aux bailleurs sociaux. La responsabilité du Gouvernement est est de faire en sorte que cet excès de liquidités soit utile à la collectivité, non seulement en finançant des projets d'intérêt public, mais aussi en servant une rémunération attractive aux épargnants. Vous mentionnez le financement de l'accélération du nucléaire par le livret A.

postale. Créé par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, ce contrat permet à La Poste de contribuer à la mission d'aménagement et de développement du territoire. Répondant au besoin vital de maintien de la présence postale dans nos territoires, il participe notamment à la mise en place des maisons de service public, comme les maisons France Services, et concourt au renforcement de l'inclusion numérique. Financé par le fonds postal national de péréquation territoriale, alimenté par un abattement de taxes locales dues par La Poste, principalement la CVAE,

Or l'article 55 de la loi de finances pour 2023 entraîne la suppression de la CVAE en deux ans, d'ici à 2024. Le Gouvernement s'est engagé à compenser cette suppression. Toutefois- les chiffres transmis le montrent -, la CVAE qui aurait été perçue en 2023,

Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Jourda, je tiens tout d'abord à réaffirmer l'engagement du Gouvernement à maintenir le soutien à La Poste pour la mise en oeuvre de cette mission de service public que constitue

Le fonds de péréquation avait ainsi pu être maintenu à son montant maximal, fixé par le contrat de présence postale à 174 millions d'euros. Pour 2023, la dotation votée en loi de finances a tenu compte de la disparition du rendement d'abattement sur la CVAE.

leurs familles et, dans certains cas, leur personnel. Désormais, pour se garer sur le parking de l'hôpital public de Nancy, au-delà des trente premières minutes gratuites, il faut débourser 6 euros pour une heure, 18 euros pour deux heures et 30 euros pour trois heures ! C'est une question importante pour le personnel de santé qui travaille dans ces hôpitaux,

pour les familles, déjà éprouvées par des situations médicales difficiles. Fort de votre expérience de médecin hospitalier, je suis certaine, monsieur le ministre, que vous êtes conscient que de nombreux patients souffrant de maladies chroniques ou en situation de handicap doivent se rendre à l'hôpital toutes les semaines, voire tous les jours, pour des soins et des traitements, et que le coût de stationnement peut devenir un frein, voire un stop à l'accès aux soins, ainsi que me l'ont rapporté de nombreux élus de mon territoire. Au cours d'une interview à BFM TV, vous avez reconnu que cette situation était problématique, tout en bottant en touche sur les solutions. Vous avez déclaré ne pas vouloir vous occuper de la question des parkings, parce que votre priorité est de redresser l'hôpital public.

Les hôpitaux publics ont le souci d'assurer la meilleure accessibilité possible pour les patients et leurs accompagnants. La gestion du stationnement ne fait pas, en elle-même, partie des missions de l'hôpital public. Les établissements peuvent donc choisir librement de confier la gestion de leur parking à des opérateurs privés.

démarche est intéressante et louable, mais sa méthode et son modèle économique et financier interrogent. En effet, le caractère obligatoire de la dépense pour les départements soulève deux problèmes.

le département doit s'engager à financer 15 % du montant de la participation de l'État, sans limitation de durée. Comme d'habitude, l'État se défausse sur les collectivités. Concrètement, selon les prévisions, pour seulement trois projets, la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) serait engagée en 2023 à hauteur de 108 000 euros pour 36 équivalents temps plein (ETP), en 2024 à hauteur de 217 000 euros pour 72 ETP

Oui, les départements souhaitent jouer leur rôle, mais sans être mobilisés auprès d'un public qui relève de l'État ! Madame la ministre, qu'envisagez-vous de faire pour ces expérimentations de « territoires zéro chômeur de longue durée » voient le jour, et cela sans faire les poches des départements ?

Vous m'interrogez sur les modalités de développement et de financement de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », issue de la loi du 14 décembre 2020. Cette expérimentation, soutenue et financée par l'État depuis la loi du 29 février 2016, a été prolongée pour une durée de cinq ans par la loi du 14 décembre 2020, afin qu'au moins cinquante territoires supplémentaires puissent être habilités, en plus des dix territoires historiques. L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État, des collectivités territoriales- en particulier les départements -, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires, ainsi que des organismes publics et privés volontaires. Dans ce cadre, l'État apporte son concours financier de différentes manières, notamment en versant la contribution au développement de l'emploi. Celle-ci correspond, pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation, à une fraction comprise entre 53 % et 102 % du Smic brut.

de 36 millions d'euros de 2022. Cela permettra le financement de 2 480 emplois au 31 décembre 2023, contre 1 120 ETP en 2022. La loi prévoit que les départements contribuent désormais de manière obligatoire, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'État. Elle prévoit également qu'un territoire ne peut être candidat à l'expérimentation que s'il a recueilli l'accord du président du conseil départemental. Il appartient au partenariat local de susciter des apports financiers complémentaires. Conformément à la loi de décembre 2020 et à son décret d'application, l'expérimentation doit faire l'objet d'une évaluation qui s'attachera à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques,

À ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, et la région Île-de-France est compétente pour l'ouverture d'un nouveau lycée dans le département du Val-d'Oise. Toutefois, l'éventuelle implantation d'un lycée dans ce secteur dépasse les limites de la seule région Île-de-France et concerne aussi la région Hauts-de-France- avec le département de l'Oise et plus particulièrement le secteur de Chaumont-en-Vexin -, mais aussi la région Normandie,

ont engagé conjointement une réflexion sur la question démographique et sur les effectifs des lycées. Cela permettra à la région d'établir des priorités quant à ses investissements et à l'État de proposer une offre scolaire adaptée. Certains territoires sont en croissance démographique démographique forte, notamment certains secteurs du Val-d'Oise, tandis que d'autres ont vu leur baisse démographique se confirmer fortement depuis plusieurs années. C'est dans ce contexte que les services de l'État et de la région expertisent les éventuels besoins de lycée dans le Vexin. Pour construire une réponse adaptée au territoire, les services des trois académies de Versailles, d'Amiens et de Normandie ont engagé un travail commun pour aboutir à un état des lieux tant du point de vue démographique que de ses incidences sur l'offre scolaire.

En se fondant sur ces analyses, les huiles essentielles pourraient être classées comme des substances chimiques, sans évaluation complète de l'ensemble des interactions entre les différents composants. Il est sans doute possible de protéger les consommateurs tout en disposant d'une parfaite connaissance scientifique des mécanismes biologiques. Je plaide pour une solution concertée, qui assure la pérennité de la production de lavande et des revenus des agriculteurs, dans des conditions optimales de sécurité des produits transformés.

C'est également dans ce cadre que nous avons porté les inquiétudes des professionnels sur la confusion possible entre perturbateurs endocriniens et substances entraînant une activité endocrinienne- cela n'est pas de même nature. L'enjeu de l'évolution de la réglementation reste l'application de la règle des mélanges à l'ensemble des substances de plus d'un constituant, dite Mocs

Première région agricole d'Europe et de France, la Nouvelle-Aquitaine souffre en effet d'une chute de près de 20 % en cinq ans du nombre de vétérinaires spécialisés en animaux de rente, et elle n'est pas la seule région dans cette situation. En second lieu, le choix d'implanter cette nouvelle école à Limoges permettrait d'ouvrir, en s'appuyant sur les facultés de médecine et de pharmacie de l'université de Limoges, un pôle de recherche unique en France dans les domaines de la médecine vétérinaire et humaine. Cette démarche s'inscrit dans la logique de la stratégie One Health, portée par la région, de manière à repenser l'approche sanitaire de la santé humaine et animale de façon globale- c'est d'autant plus utile au regard de la récente pandémie. Il s'agit d'organiser un écosystème fédérant les praticiens vétérinaires, les formations universitaires, les laboratoires de recherche et les entreprises leaders du secteur. La future école vétérinaire serait innovante à plus d'un titre : : école publique avec classe préparatoire intégrée aux cinq années d'études, recrutement drainant de nouveaux profils issus du monde agricole et rural, approche pédagogique innovante ouverte sur la pratique. La région Nouvelle-Aquitaine est prête à financer une partie de l'implantation de la nouvelle école, mais a naturellement besoin du soutien de l'État pour concrétiser ce projet. Or, à ce jour, aucune avancée n'a été obtenue, et le projet semble, hélas, au point mort. L'État entend-il s'engager clairement dans ce projet essentiel pour la Haute-Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine ?

où les études sont plus courtes et moins onéreuses. Pour le premier pays agricole d'Europe, convenez que c'est une problématique majeure, qui aura, et qui a même déjà, des conséquences sur l'avenir de l'élevage dans les territoires. Lorsque les collectivités locales proposent un projet innovant, l'État doit répondre présent pour les soutenir.

ne relève pas tout à fait de mon périmètre. Cette indexation permet de faire évoluer, au cours de la durée de vie du contrat d'achat ou de complément de rémunération, le tarif pour l'électricité pour l'électricité produite par l'installation. Ce tarif est initialement fixé par contrat entre EDF Obligation d'achat (EDF OA), cocontractant, et l'exploitant du parc photovoltaïque. Le loyer versé à l'agriculteur par l'exploitant du parc est donc bien fixé par un contrat entre personnes privées, ainsi que vous l'avez rappelé, et il ne dépend dépend pas directement du niveau du tarif dont bénéficie l'exploitant du parc photovoltaïque. Je tiens aussi à rappeler que l'État apporte un complément de rémunération par rapport au prix de marché pour garantir l'équilibre des projets. Il n'est donc pas illégitime que nous intervenions dans les dans les conditions de mise en oeuvre des contrats. Je réponds ainsi à votre question de principe. Néanmoins, face aux difficultés que les porteurs de projets ont pu connaître ces derniers mois, des mesures d'urgence ont été mises en place par le ministère de la transition énergétique, dont la prise en compte de l'augmentation des coûts des matières premières pour les panneaux photovoltaïques, dans une formule d'indexation du tarif avant activation du contrat. Par la prise en compte de ces différents éléments dans les tarifs d'achat de l'électricité produite, le Gouvernement souhaite renforcer la résilience des projets photovoltaïques bénéficiant de contrats d'achat de l'électricité produite ou de complément de rémunération, afin de minimiser les risques et les externalités négatives sur les parties tierces à l'opération- dont l'agriculteur dans le cas d'une opération d'agrivoltaïsme. Cette indexation pourra toutefois être appelée à évoluer Cette indexation pourra toutefois être appelée à évoluer en fonction des discussions à venir sur l'agrivoltaïsme, pour que la formule reflète mieux la réalité des projets, si tel n'était déjà pas le cas aujourd'hui.